rectifié. L'article 19 a été inséré par la commission, en vue de supprimer la reprise automatique du droit de préemption urbain par le préfet, lorsque la carence d'une commune est prononcée.

Mélot, tend à réinstaurer la reprise du droit de préemption urbain par le préfet, tout en supprimant son caractère automatique. Il s'agit de pouvoir cibler les communes concernées et, ainsi, d'améliorer l'action de l'État en la matière et l'efficience de cet outil, notamment lorsqu'il est possible de le déléguer à un EPF ou à un bailleur social.

à modifier le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, afin de réinstaurer la reprise du droit de préemption urbain par le préfet, tout en supprimant son caractère automatique.

La procédure doit ensuite permettre de saisir la commission nationale, qui peut, elle, décider de recommander au ministre chargé du logement un aménagement des obligations prévues

Il me paraît juste irrationnel, pour rester sympathique, de se priver de cette procédure, car il n'y a plus, du coup, aucun moyen légal de réduire l'objectif impératif.

départementales n'auront plus de raison d'être du fait de la création du contrat de mixité sociale. Quant à la commission nationale SRU, elle reste bien évidemment compétente pour le bilan

de logements concerné. L'objectif est d'assurer la cohérence entre les orientations des politiques locales de l'habitat, décidées par les collectivités, et les stratégies propres de chacun des bailleurs présents sur le territoire.

n° 1590 rectifié . Les politiques locales de l'habitat sont avant tout des politiques partenariales. Les organismes de logement social interviennent aux côtés des collectivités pour répondre aux besoins de logements nouveaux, satisfaire les obligations en matière de mixité sociale et conduire les politiques de peuplement. Les collectivités locales contribuent activement à la production du parc social et à son évolution, en apportant des aides directes ou indirectes. Il semble donc logique qu'elles soient étroitement associées à l'évolution du patrimoine des organismes de logement social pour le parc se situant sur leur territoire. Cet amendement vise à ce que soit établie par les collectivités,

que la convention soit annexée au PLH et qu'elle détermine, en fonction des orientations de celui-ci pour chacun des organismes de logement social signataires, la stratégie patrimoniale à déployer sur le territoire.

les politiques de loyer et leur évolution et la gestion du parc en termes de services rendus. L'objectif est d'assurer une cohérence complète en matière de logement social à l'échelle d'un territoire entre les orientations des politiques locales

La production de logements locatifs intermédiaires est soumise non plus à un agrément de l'État, mais à une simple déclaration. Or de nombreuses communes déficitaires dans le cadre de la loi SRU continuent à produire des logements locatifs intermédiaires au détriment du logement locatif social.

rétablirait une assimilation entre logements locatifs intermédiaires et logements locatifs sociaux. Or les logements intermédiaires ne sont pas des logements sociaux

des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) sur les garanties d'emprunt qui sont accordées par les collectivités territoriales aux organismes de foncier solidaire (OFS). Les OFS demandent que leurs emprunts puissent être garantis par les départements et par les régions

en cohérence avec le nouveau partage des responsabilités dans ce domaine, notamment celles confiées aux collectivités locales au titre de la délégation des aides à la pierre. Il est proposé de faire évoluer les missions des CRHH autour de feuilles de route claires et de responsabilités renforcées dans une déclinaison locale des dispositifs nationaux en faveur de l'habitat. À ce titre, pour isoler la vocation consultative des CRHH, largement ouverte aux différentes parties prenantes des politiques du logement, et pour une capacité qui se rapprocherait davantage de prises de décision concernant plus directement les acteurs locaux financeurs des politiques du logement, nous suggérons de créer au sein des CRHH un comité des financeurs. Celui-ci aurait vocation à regrouper, entre autres, les services déconcentrés de l'État,

à terme des « PLUiH » dans tous les territoires. Donner un caractère plus opérationnel à la dimension régionale de la politique du logement et de l'habitat, c'est aussi mettre en cohérence les moyens et les objectifs que l'on veut se fixer.

Toute opération d'aménagement qui a reçu des subsides publics doit participer à l'effort national de construction de logements abordables, ce pour garantir le droit au logement pour tous, constitutionnellement

d'aider les bailleurs sociaux à construire et à développer l'offre dans les communes rurales. L'enveloppe du plan de relance sur la réhabilitation des logements sociaux va permettre à ces bailleurs d'entreprendre les travaux de rénovation nécessaires.

urbaines et industrielles soient conditionnées, lorsque les terrains dépollués ont pour destination la construction de logements, à la fixation d'un pourcentage minimum de logements sociaux ou de logements éligibles à l'accession sociale à la propriété.

les communes investissent beaucoup et se mobilisent. Concernant le logement, nous avons tous été confrontés dans nos fonctions respectives à des concitoyens en recherche d'informations pour engager des travaux de rénovation de leur logement.

d'un collège des représentants des collectivités territoriales, d'un collège des représentants des professionnels du logement et de l'immobilier et d'un collège des représentants d'organismes qui interviennent dans le domaine de l'accueil, du soutien et de l'hébergement. Le règlement du

peut mener des expérimentations ou des adaptations des règles nationales et participer à leur évaluation. Nous proposons de renforcer encore la mission de concertation et de pilotage du CRHH, notamment en matière de maîtrise des coûts des opérations de construction.

La part de la VEFA dans la production de logements sociaux a été multipliée par douze en dix ans ; les valeurs foncières et les prix de la VEFA ne cessent d'augmenter. Cet outil reste néanmoins incontournable pour la construction de logements sociaux en zone tendue, d'où la nécessité d'encadrer les prix sur un territoire donné. Cette mission pourrait utilement être confiée au CRHH. Quel est l'avis

tels dispositifs permettent aux élus locaux de lutter contre l'explosion du prix des logements neufs. Cet effort nous paraît essentiel, car il permet d'agir sur le foncier privé et de contrecarrer la spéculation

pour les baux conclus postérieurement au 1 janvier 2023. Selon nous, une telle mesure n'est pas opportune : elle conduirait à imposer à des ménages modestes la location d'une place de stationnement, y compris lorsqu'ils ne possèdent pas de véhicule. Aussi, nous proposons la suppression de cet article.

notamment dans la ville dense. Aussi, je suis favorable à ces amendements de suppression.

PLU. Destinée à optimiser la gestion des résidences d'HLM, cette dissociation est devenue un véritable obstacle pour les élus et les populations. Elle nuit à l'acceptabilité du logement social, car elle conduit à l'encombrement de la voirie communale et pose des problèmes de sécurité.

pour ne pas empêcher une appréciation locale et différenciée, en fonction des communes concernées, quand bien même elles dénombreraient plus de 40 % de logements sociaux. Mais c'est aussi le rôle de la loi que d'affirmer un certain nombre de règles générales. En l'occurrence, nous voulons voir instaurer cette loi SRU

au titre du droit au logement opposable issu de la loi DALO et aux publics prioritaires s'appliquera uniformément pour chaque bailleur social. Cette disposition est de nature à fragiliser les conventions intercommunales d'attribution,

et à reporter de deux ans les réformes de la gestion en flux des réservations et de la cotation des demandes de logements sociaux. Comme l'indique le rapport, la commission a estimé nécessaire de tirer les conséquences de la crise sanitaire et de prendre en compte le besoin de logements

la cotation de la demande et de la gestion en flux des réservations de logements sociaux étant reportée à la fin de l'année 2023, cet amendement tend à prolonger de deux ans le calendrier fixé pour conclure les CIA,

Il s'agit de dispositions anciennes, qui laissaient déjà du temps aux intercommunalités pour élaborer leurs conventions intercommunales d'attribution ; il est vraiment nécessaire d'accélérer, sinon nous n'atteindrons jamais nos objectifs de mixité sociale.

Y a-t-il un quelconque intérêt à ajouter une énième catégorie de personnes prioritaires, alors que les demandeurs sont de plus en plus nombreux et que l'attribution des logements est en baisse en raison d'une plus faible rotation que par le passé ? Est-il souhaitable de mettre en concurrence des personnes sans logement et ces travailleurs clés ? Par ailleurs, est-il bienvenu de consacrer législativement une dualité entre ceux qui exerceraient un métier essentiel et les autres ? À ces interrogations, nous vous répondons par la négative.

ils appellent aussi à l'intervention étatique la production de logements pour répondre à la demande exponentielle. En somme, ce nouveau critère ne ferait qu'aggraver une situation déjà difficile. Quel M. Max Brisson. Les objectifs purement comptables et administratifs reviennent, ces dernières années, à écarter les habitants pourtant éligibles de l'accès au logement social de leur propre commune.

parce que la crise sanitaire a vraiment démontré le caractère essentiel de certaines activités pour la continuité de la vie de la Nation. La notion de « travailleur clé » ne porte pas un jugement de valeur sur un métier plus ou moins essentiel, mais souligne que certaines missions doivent être assurées de façon continue et ne peuvent pas

? Cet amendement a déjà été discuté en commission et a reçu un avis défavorable, car il va à l'encontre d'un principe essentiel d'attribution des logements sociaux. Si le lien avec la commune ne peut être négligé, notamment sur le plan familial, l'attribution de logements sociaux implique également l'accueil de nouvelles populations, en particulier parmi les publics prioritaires en difficulté. J'en demande donc le

rectifié, quant à lui, tend à ce que les objectifs légaux d'attribution soient respectés pour pallier le mal-logement des demandeurs les plus modestes, une fois de plus. Il vise en particulier les personnes prioritaires et reconnues au titre du DALO par les bailleurs sociaux.

qui sont encore trop peu nombreuses. J'ai cité les chiffres de l'étude d'impact d'octobre 2020, qui fait état de très peu de conventions intercommunales d'attribution signées. Il faut prendre des mesures pour pallier leur absence. Nous sommes en accord avec cette approche réaliste et donc défavorables à ces amendements.

Le niveau du premier quartile est défini annuellement par arrêté et il nous semble que cet indicateur n'est pas suffisamment pertinent, sans compter ses effets de seuil.

vous proposez de préciser et de compléter la liste des publics prioritaires pour l'attribution de logements sociaux au niveau local. Nous sommes nombreux à réfléchir à cet objectif, mais votre proposition me paraît dangereuse à mettre en oeuvre

Cet amendement vise à introduire une exception à la gestion en flux au profit des établissements de santé, car ceux-ci ont fait construire des logements sociaux sur leur domaine privé, à proximité immédiate des lieux de travail. L'application de la gestion en flux à ces logements pourrait réduire à néant l'effort accompli depuis plusieurs années pour loger ces travailleurs essentiels à proximité de leur lieu de travail. Cet amendement s'inscrit donc pleinement dans l'objectif de ce projet de loi. Nous partageons la volonté de reconnaître le rôle déterminant

n° 80 rectifié. La loi fixe des objectifs d'attribution visant à mettre en oeuvre le droit au logement et à favoriser l'équilibre social et la mixité des villes et des quartiers.

Pour rendre cet objectif opérationnel, celui-ci doit également être mis en oeuvre par les réservataires chargés de la désignation des candidats. Cet amendement vise à clarifier le fait

353-15 du code de la construction et de l'habitation, en cas de démolition, le bailleur est tenu de faire au maximum trois offres de relogement correspondant aux besoins personnels ou familiaux des occupants, dans le respect des dispositions de l'article 13 de la loi du 1 septembre 1948. Le présent amendement a pour objet de préciser le rôle de la commission d'attribution et d'examen de l'occupation des logements, qui est plus limité en ce cas. Il apparaît néanmoins nécessaire qu'elle soit informée de ces relogements après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants, ainsi que de l'offre de relogement ayant fait l'objet d'une acceptation.

Il favorise tout particulièrement la pleine intégration de ces quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant notamment leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale. Afin de compléter les leviers actuellement mobilisables pour augmenter la diversité de l'habitat et favoriser la mixité fonctionnelle dans les quartiers concernés par le NPNRU, qui constituent des objectifs fondamentaux du programme, cet article propose de créer une nouvelle disposition pour permettre le changement de statut résidentiel- accession, locatif libre -ou d'usage d'immeubles de logements locatifs sociaux par la vente de tout ou partie de ces bâtiments. Le dispositif encadre les conditions de réalisation de ces opérations, ainsi que l'évolution nécessaire du droit au maintien dans les lieux pour les permettre. de ne pas générer de potentielles ventes au profit de marchands de sommeil, il est précisé que celui-ci ne s'applique qu'aux ventes en bloc d'au moins cinq logements à des personnes morales. Compte tenu de l'obligation de respect du taux SRU, la vente n'est pas permise dans les communes qui, concernées par l'obligation d'atteindre 20 % ou 25 % de logements sociaux, ne les atteindraient pas. Cette nouvelle disposition participera à l'amplification et à l'accélération du nouveau programme national de renouvellement urbain. Elle favorisera l'accélération de la diversification résidentielle ou fonctionnelle dans les quartiers du et réduira l'impact financier et environnemental des projets en offrant une alternative à la démolition des immeubles. Elle contribuera également aux politiques de rééquilibrage de l'offre résidentielle en visant la reconstruction de l'offre de logements locatifs sociaux ainsi diminuée à l'extérieur des QPV.

dans les programmes de renouvellement urbain en cas de démolition d'immeuble, rien n'est prévu lorsque l'on décide de conserver un immeuble, mais de l'évacuer en vue d'un changement complet d'usage

Lorsqu'il est plus facile de faire valoir ses droits, le non-recours diminue et l'effectivité du droit progresse. Mieux assurer les droits des personnes est un enjeu fondamental et atteignable

vise à professionnaliser les commissions de médiation. Il prévoit ainsi que la présidence en soit exercée par un magistrat, en exercice ou honoraire, ou par une personnalité qualifiée en droit. L'objectif est, d'une part, d'améliorer la sécurité juridique des décisions,

Une telle modification de leur composition aurait sans nul doute un effet positif sur la qualité rédactionnelle des décisions rendues, améliorant de fait la sécurité juridique de ces dernières. Vous conviendrez que cela permettrait de plus de parer au risque de recours pour excès de pouvoir, notamment, mais aussi et surtout à la menace des sanctions qui peuvent en

» me semble beaucoup trop imprécise. Par ailleurs, compte tenu de la charge de travail des magistrats, je doute qu'il soit pertinent de leur confier une mission complémentaire. Avis défavorable. Quel est

La réglementation prévoit que ces commissions sont présidées par une personnalité qualifiée désignée par le préfet de département. Dans ce cadre, ce dernier peut désigner une personnalité qualifiée en droit.

Lorsque le juge administratif statue favorablement sur le recours en injonction de relogement d'un ménage reconnu au titre du DALO qui n'a pas obtenu de proposition de logement dans les délais légaux, l'État est condamné à verser une astreinte. Aujourd'hui, celle-ci est intégralement versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, un programme créé en 2011 dans le but de financer l'accompagnement personnalisé de ménages prioritaires. Le fonctionnement de ce fonds pose deux difficultés majeures. Tout d'abord, on ne peut se satisfaire

Il apparaît dès lors indispensable d'opérer une refonte des modalités de versement de cette astreinte en la répartissant équitablement entre le Fonds national précité et le requérant.

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a institué, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans, un dispositif dérogatoire autorisant le gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année, à louer les locaux inoccupés pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1 septembre, et ce particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l'État. Cet amendement a pour objet de rendre ce dispositif pérenne en l'insérant dans le code de la

soit facultatif et qu'il soit mis en place sur l'initiative de l'établissement public de coopération intercommunale.

un outil d'aide à la décision objectif et transparent permettant de départager plusieurs demandes pour un même logement. Il s'impose à tous les EPCI tenus de se doter d'un programme local de l'habitat ou ayant la compétence habitat et au moins un QPV. Toutefois, les territoires situés en zone détendue ne sont pas concernés par un déséquilibre entre l'offre et la demande. Dans un objectif de territorialisation des politiques de l'habitat, nous proposons par cet amendement que dans ces territoires, ce dispositif de cotation soit facultatif et qu'il soit mis en place sur l'initiative de l'EPCI.

titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi et afin de résorber de manière significative la vacance anormalement longue affectant les logements locatifs sociaux, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence habitat dans les zones géographiques B2 et C, qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande, puissent déroger aux règles d'attribution. Le recours à la cotation et à la gestion en flux en matière d'attribution serait donc laissé à l'appréciation du ou des établissements publics volontaires. En outre, dans le cadre de cette expérimentation, les établissements publics volontaires pourront procéder à des changements d'usage de logement, nonobstant les clauses et conditions de la convention mentionnée de l'article L. 831 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il est avéré que cela permet de répondre à des besoins en matière de logement

Mme Nassimah Dindar. Durant la crise sanitaire, il a été permis aux bailleurs sociaux de déroger aux dispositions de l'article L. 441-2

Cette mesure ne nous semble pas utile, car le maire de la commune, en lien avec l'EPCI, joue déjà un rôle essentiel dans la stratégie d'attribution de sa commune : il est membre de la Caleol et dispose d'une voix prépondérante. Par ailleurs, le parc social non réservé des bailleurs sociaux est très utile pour gérer les mutations ou les relogements nécessités par les opérations de réhabilitation ou de lutte contre l'habitat indigne. Enfin, les droits de réservation sont une composante significative du financement des opérations de logement social, déjà mis à mal par les mesures prises par le Gouvernement ces dernières années. Aussi notre amendement propose-t-il de supprimer cet article.

non réservés dont sont titulaires les bailleurs sociaux, déduction faite de ceux qui sont repris par le préfet, lorsque les bailleurs sociaux ne respectent pas leurs objectifs d'attribution au bénéfice des ménages prioritaires, dont les DALO. Le financement des droits de réservation, et donc la constitution de ces contingents, est une composante importante du modèle de financement des organismes HLM. En effet, la part des logements réservés dans le cadre d'une convention de réservation en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts par les communes peut représenter globalement jusqu'à 20 % du flux annuel sur le territoire d'une commune. Des réservations complémentaires peuvent être obtenues en contrepartie du financement d'un apport de terrain. Le transfert de logements non réservés vers le contingent communal, l'article 22 , constitue une remise en cause des mécanismes précités. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est prévu pour le préfet, qui reprend l'exercice d'attribution pour un tour au bénéfice des ménages prioritaires, l'article 22 ne prévoit pas une telle

Salmon, pour présenter l'amendement n° 1208. En faisant du maire l'autorité d'attribution par défaut des logements non réservés, l'article 22 pourrait nuire à la transparence et à l'égalité des chances des demandeurs. En attestent plusieurs rapports de l'Agence nationale de contrôle du logement social qui ont souligné les potentielles dérives pouvant résulter d'un monopole de la concentration de l'attribution des logements sociaux dans les mains des maires. Une telle mesure serait d'autant plus malvenue que la procédure actuelle est satisfaisante, notamment parce qu'elle garantit la représentativité des élus locaux dans les conseils d'administration des organismes HLM.

rectifié. Le financement des droits de réservation, et donc la constitution des contingents, est une composante importante du modèle de financement des organismes de logement social. En prévoyant un transfert des logements non réservés vers le contingent communal, l'article 22 constitue une remise en cause importante des mécanismes précités. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est prévu pour le préfet, qui reprend l'exercice d'attribution pour un tour au bénéfice des ménages prioritaires, l'article 22 ne prévoit pas une telle affectation des logements repris par les communes, ce qui prive ce transfert de

pour un tour, le transfert prévu par la commission est un transfert définitif des capacités d'attribution. Deuxièmement, lorsque le préfet reprend l'exercice du droit d'attribution des logements non réservés, il procède aux attributions au bénéfice unique des ménages prioritaires,

Ce nouvel article ouvre en outre la possibilité de refuser l'attribution d'un logement dans une résidence à enjeu prioritaire à un ménage dont la candidature serait susceptible d'accentuer la fragilité sociale de la résidence. Notre amendement a pour objet de supprimer ces nouvelles dispositions, car la vocation du parc social est d'apporter des solutions de logement aux personnes de ressources modestes et aux personnes défavorisées, en contribuant à l'équilibre social et donc à la cohésion des territoires les plus fragiles. ailleurs, il revient aux conférences intercommunales du logement de définir les résidences ou secteurs à enjeu de mixité, ainsi que les publics à orienter en priorité sur ces résidences.

que nous avons voulu mettre en oeuvre afin de continuer à casser les ghettos. Nous avons tous l'expérience, dans nos communes, de ménages en difficulté qui se voient, en réalité, très souvent attribuer des logements dans des résidences déjà fragiles. De fait, les loyers y sont moins chers,

comme Grenoble et vingt-sept communes environnantes, Montpellier, Lyon, Bordeaux, Villeurbanne, Est Ensemble, Plaine Commune et onze communes du Grand-Orly Seine Bièvre. L'encadrement des loyers, là où il a été appliqué, s'est révélé particulièrement efficace. En deux ans, à Paris, il a permis de diminuer le nombre et le niveau des compléments de loyers supérieurs aux loyers plafonds imposés par quartier et par type de logement. La part des dépassements est en effet passée de 26 % en 2015 à 23 % en 2016

l'amendement n° 485. Le projet de loi prolonge le dispositif expérimental de l'encadrement des loyers jusqu'au 23 novembre 2026. À ce jour, une dizaine de candidatures ont été déposées pour participer à l'expérimentation. de permettre une évaluation sur un périmètre plus étendu, notre amendement tend à rouvrir la période pendant laquelle les intercommunalités compétentes et collectivités éligibles, situées en zone tendue, peuvent déposer une candidature pour mettre en oeuvre le dispositif expérimental d'encadrement des loyers sur leur territoire. Cette période de candidature s'est achevée le 23 novembre 2020. Il est donc proposé d'autoriser de nouvelles candidatures jusqu'au 23 novembre 2022.

Or personne n'ignore que, en raison du contexte sanitaire et économique pour le moins inédit que nous connaissons depuis maintenant plus d'un an, de nombreuses communes n'ont pas pu déposer à temps leur candidature pour bénéficier de ce dispositif. De plus, si l'on veut mesurer l'efficacité réelle de cette mesure, il est nécessaire de permettre à davantage de communes d'en bénéficier. Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons de prolonger de deux ans ladite période de candidature, soit jusqu'au 23 novembre 2022.

la période pendant laquelle les intercommunalités compétentes et collectivités à statut particulier, situées en zone tendue, peuvent déposer une candidature visant à proposer la mise en oeuvre sur leur territoire du dispositif expérimental d'encadrement des loyers. Quel est l'avis de la commission des affaires

en matière de politique publique comme « le recours à une méthode consistant à mettre temporairement en oeuvre un dispositif afin, par une évaluation rigoureuse, d'en mesurer les effets, au regard des objectifs poursuivis ».

mais j'ajoute que ce comité de pilotage pourra être institué pour chaque territoire afin de garantir surtout le partage de l'information et des analyses et, le cas échéant, l'adaptation des conditions de mise en oeuvre du dispositif. Ces travaux permettraient d'alimenter utilement l'évaluation nationale du dispositif qui, bien sûr, doit être menée.

précédents, le présent amendement vise à améliorer le dispositif d'évaluation de l'expérimentation de l'encadrement des loyers, en y associant mieux les collectivités par le biais d'une instance de suivi au niveau local. Je me permets de rappeler que la mise en oeuvre de cette expérimentation est l'expression du volontarisme des collectivités territoriales, car ce sont elles qui en ont fait la demande afin de prendre en main leur politique du logement et de l'habitat, notamment à des fins de maintien de la mixité sociale. En outre, personne ne peut nier l'implication des collectivités dans la réussite de cette expérimentation. Elles ont en effet mobilisé leurs services, leurs moyens pour l'accès à l'information et à la communication, le financement de la collecte des données, entre Or, à ce jour, le dispositif ne prévoit pas l'association des collectivités territoriales dans le suivi et l'évaluation du dispositif en vue de sa pérennisation. C'est la raison pour laquelle le présent amendement a pour objet que l'évaluation soit menée par un comité associant l'État, les collectivités participantes et les acteurs centraux de la politique du logement. Il vise également à ce que, pour chaque territoire, un comité de pilotage soit institué, afin de garantir le partage de l'information et des analyses et, le cas échéant, l'adaptation des conditions de mise en oeuvre du dispositif.

ne paraissent pas nécessaires au regard de la manière dont sont menées les évaluations des expérimentations. Par exemple, concernant les courts séjours en résidence universitaire que nous avons évoqués précédemment, l'administration a de fait procédé

vise à adapter le système d'encadrement des loyers en fixant le loyer de référence majoré à 10 % au lieu de 20 % en Île-de-France, région où les loyers sont les plus élevés, ce qui rend l'accès au parc locatif privé très difficile pour de nombreux ménages. ménages. En effet, si l'on considère les chiffres de 2019, les écarts de prix entre les logements à Paris et en banlieue sont les plus importants que l'on puisse observer dans l'ensemble du territoire français. Ainsi, en prenant le prix médian au mètre carré, les chiffres sont éloquents de 16 à 31 euros mensuels le mètre carré loué dans la capitale, et de 13 à 19 euros dans le reste des communes franciliennes. En 2015, l'Insee relevait d'ailleurs que les prix en région parisienne dépassaient de 9

que le législateur ne pouvait porter atteinte au droit de propriété que dans des conditions strictes et limitées. Il a jugé que le dispositif d'encadrement des loyers implique

qui déterminent habituellement le montant du loyer. J'ajoute que le Conseil constitutionnel s'est opposé au dispositif qui prévoyait que le montant du loyer de référence majoré et le montant du loyer de référence minoré seraient fixés non pas respectivement à plus 20 % et moins 30 % du loyer de référence, mais à l'intérieur de ces limites. L'avis est donc défavorable.

tant pour les propriétaires que pour les locataires. Dans certains territoires, les commissions départementales de conciliation soulignent une augmentation notable des saisines relatives à la contestation du complément de loyer. Ce dernier peut en effet être utilisé par les propriétaires pour atteindre un niveau de loyer supérieur qui est permis dans le cadre du dispositif d'encadrement des loyers, hors charges, tout en paraissant respecter le loyer de référence majoré. Dans ce contexte, il est proposé de compléter la définition en s'inspirant d'exemples rencontrés sur le terrain, notamment concernant l'existence d'équipements ou de matériaux luxueux, d'un extérieur comme une terrasse ou un jardin, d'un espace complémentaire comme un parking, une grande cave ou un sous-sol, ou de toute aménité particulière liée au logement et qui le distingue de ceux de même catégorie qui sont situés dans le même secteur géographique. secteur géographique. La précision de la définition du complément de loyer permettra d'accompagner aussi bien les propriétaires de bonne foi, qui s'interrogent sur les éléments pouvant donner lieu à un complément,

à ces trois amendements, car ils sont contraires à la jurisprudence du Conseil constitutionnel que je viens de citer. En effet, celui-ci a déclaré contraires à la Constitution les dispositions qui réservaient la possibilité d'un complément de loyer à des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et leur ampleur. Le législateur ne saurait interdire que d'autres caractéristiques qui sont déterminantes pour la fixation du loyer

Ainsi, sur les 17 000 annonces locatives passées au crible durant ces douze derniers mois, une annonce immobilière sur deux, précisément

Si l'on veut véritablement contenir la hausse des loyers, éviter des augmentations excessives dans des territoires au marché locatif privé particulièrement tendu, préserver ainsi l'accès au logement des ménages de la classe moyenne, contribuer au maintien de la mixité sociale en zone tendue, il est nécessaire de mieux faire respecter la loi. Il faut pour cela que le montant de l'amende administrative encourue en cas de non-respect de l'encadrement des loyers soit véritablement dissuasif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pourquoi nous proposons de doubler chacun des deux plafonds des amendes encourues, soit une évolution de 5 000 à 10 000 euros pour les personnes physiques et de 15 000 à 30 000 euros pour les personnes morales.

Mme la ministre.

Si nous pouvons le faire dans une ville comme Paris, vous en constaterez les effets extrêmement bénéfiques, notamment pour les couches sociales moyennes, qui sont obligées de quitter la capitale à cause d'une spéculation immobilière effrénée dans certains secteurs tendus. Je mets

Avec cet amendement, nous souhaitons clarifier les alinéas 2 et 3 portant modification des articles 206 et 209 de ladite loi. En effet, ces articles consacrent les notions de lots transitoires et de parties communes spéciales, ainsi que celle de jouissance privative, en imposant leur mention au règlement de copropriété. Ces dispositions, censées être des mesures transitoires, sont sources de difficultés d'interprétation et sont comprises par la doctrine majoritaire comme remettant en cause les droits des copropriétaires concernés, faute de mise en conformité des règlements de copropriété dans les délais impartis. Pour éviter toute nouvelle difficulté d'interprétation, le présent amendement vise à préciser que cette mention est sans incidence sur l'existence de ces lots et parties communes. Quel

Cet article vise à harmoniser les régimes de délégation de compétences de l'État aux intercommunalités et métropoles en matière de logement social et d'hébergement. Cette nouvelle rédaction contenue dans le PJL nous laisse extrêmement dubitatifs sur ses possibilités, notamment en ce qui concerne les compétences régaliennes de l'État en matière d'hébergement et de droit au logement opposable (DALO). Apparemment, selon l'étude d'impact, en 2020, moins de 4 % des délégataires avaient inclus dans la convention de délégation les compétences en matière de gestion du DALO et de réservation de logements sociaux. Par ailleurs, aucune convention ne portait sur les compétences relatives à la veille sociale, l'accueil et l'hébergement d'urgence. Nous estimons donc qu'en lieu et place d'une réécriture du code général des collectivités territoriales et du code de la construction pour apporter de la souplesse dans ces délégations de compétences, il eût été plus opportun de revoir l'ensemble de ces délégations pour étudier l'opportunité de leur maintien. Telle est la raison de cette demande de suppression. L'amendement n° 1348 n'est pas soutenu. Quel est l'avis de la commission

satisfait en droit, car le système de délégation prévoit, par définition, que les compétences sont exercées au nom et pour le compte du délégant, en l'occurrence l'État. À l'inverse, l'introduction d'une telle mention

Sassone. Il s'agit de rétablir les deux délégations, parce qu'il me semble que c'est par erreur que l'article 25 a abrogé la possibilité pour les métropoles de demander la délégation des agréments d'aliénation des logements sociaux à travers les conventions d'utilité sociale, les CUS. Le projet de loi de décentralisation et de différenciation ne peut conduire

supprimé la possibilité de déléguer la délivrance des agréments de vente HLM aux bailleurs sociaux. Je suis donc favorable à votre proposition. Le Gouvernement propose toutefois un sous-amendement de coordination,

Le présent amendement vise à supprimer l'ajout dans la loi d'une disposition déjà codifiée. En effet, les départements peuvent déjà bénéficier d'une délégation de compétences de l'État de l'État en matière d'aides à la pierre, aux termes de l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation. Cette disposition présente de plus un risque de

privé. De nombreuses intercommunalités ont saisi cette possibilité et sont devenues délégataires des aides à la pierre. La lutte contre la précarité énergétique des logements est aujourd'hui un enjeu central des ambitions du Gouvernement en matière de transition écologique. De nombreux dispositifs d'aide ont vu le jour, notamment, depuis 2020, le dispositif MaPrimeRenov', en remplacement du (CITE). Ce dispositif, qui connaît un important succès, dispose d'une enveloppe financière qui a été fortement bonifiée dans le cadre du plan France Relance. Il a été étendu à l'ensemble des propriétaires et copropriétés. Actuellement, MaPrimeRénov's'appuie sur un pilotage national, et le lien avec les priorités des politiques menées localement par les collectivités n'est pas assuré. Le présent amendement, porté par Fabien Genet, vise à permettre aux intercommunalités délégataires des aides à la pierre de pouvoir gérer directement les crédits correspondant aux aides accordées sur leur territoire.

qui accorde aujourd'hui MaPrimeRenov', au profit d'acteurs locaux, quand bien même il s'agirait d'intercommunalités. Cela introduirait beaucoup de complexité et réduirait, de fait, la visibilité et la capacité de mesurer les effets des politiques menées, alors que nous devons tous faire

est ainsi libellé : La parole est à M. Loïc Hervé. Cet amendement vise à amplifier le mouvement de territorialisation des politiques de l'habitat engagé depuis de nombreuses années avec l'essor des programmes locaux de l'habitat, les délégations des aides à la pierre, les plans de gestion de la demande et le partenariat quotidien avec les opérateurs. repenser les modalités de mise en oeuvre des orientations nationales à travers une nouvelle contractualisation beaucoup plus ambitieuse entre l'État et les autorités organisatrices, permettant des expérimentations nouvelles et des capacités d'ajustement des seuils ou ou zonages nationaux aux réalités locales. Nous souhaitons enfin assurer la participation active des collectivités au processus de recomposition du tissu des organismes de logements sociaux dans un souci de préservation de son ancrage dans les bassins de vie et les réalités locales. Quel est l'avis de la commission des ? Je suis personnellement favorable au principe, car j'estime que l'intercommunalité est véritablement le bon niveau pour déployer les politiques locales de l'habitat. C'est déjà le cas pour un certain nombre de dispositifs. À mon avis, c'est l'évolution que nous devrons suivre dans les prochaines années. Pour autant, j'ai conscience que cet amendement très important arrive en fin de discussion de la partie « logement » du texte, qui a focalisé l'attention sur beaucoup d'autres sujets, et ce sans avoir fait l'objet de toutes les consultations juridiques et concertations nécessaires avec les associations d'élus.

de la définition et de la mise en oeuvre de toutes les politiques locales de l'habitat sur le territoire. Cependant, la notion d'autorité organisatrice crée un nouveau concept, qui vient s'ajouter à ceux, déjà bien établis dans notre droit,

un peu flou, si je puis dire. Le Gouvernement a connaissance de ce projet, qui a été défendu notamment par qu'il nécessite encore des discussions. À mon sens, l'État doit conserver certaines compétences pour garantir l'équité entre les territoires, en tenant compte des spécificités de chacun. Des transferts supplémentaires portant sur la révision des zonages liés aux dispositifs d'investissement locatif et de prêt à taux zéro ou sur l'attribution des aides MaPrimeRénov'ne sont pas souhaitables, car ils nuiraient à la nécessaire cohérence de ces politiques au niveau national.

la prochaine séance. Mes chers collègues, je vous informe que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique